La séance est reprise. Nous poursuivons l'examen du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d'orientation des mobilités.

loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a tout d'abord étendu aux piétons le bénéfice de ladite servitude, avec pour effet de modifier sa vocation d'origine en prévoyant une possibilité d'accès aux berges des cours d'eau assortie d'aucune dérogation ni souplesse, créant ainsi une difficulté à la fois pratique et juridique, puisque les berges ne sont pas aménagées en ce sens. sens. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l'emprise de la servitude, afin d'assurer le cheminement continu de piétons. Dans les faits, cette loi peine à s'appliquer et présente des effets indésirables, tant pour la sécurité des piétons que pour la préservation des espaces naturels. Le présent amendement, en tendant à clarifier la priorité dans la superposition des servitudes, vise une solution qui maintient l'extension faite aux piétons en 2006 tout en ménageant les zones classées et/ou inscrites. Dans ces zones sensibles, l'autorité administrative compétente pourra favoriser le déploiement des voies vertes, qui ont déjà été réalisées avec succès par de nombreuses collectivités en mettant en place des conventions de passage avec les propriétaires riverains à l'issue d'échanges concertés.

Deux rapports du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, diligentés par le ministère chargé du développement durable et des transports, ont mis en évidence les difficultés, voire les impossibilités d'application de la loi. loi. Cet amendement, en comportant une alternative pour assurer la continuité du cheminement, vise à résoudre de nombreuses situations de blocage préalablement constatées.

peut apporter des solutions intéressantes en matière d'aménagement, d'entretien et de valorisation des lieux, mais que cela suppose en revanche une adaptation de la gouvernance existante. Il faudrait donc plutôt prévoir d'élargir la concertation au moment de la définition de ces plans départementaux aux chambres d'agriculture et aux associations des propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux.

rectifié. Le présent amendement tend à créer une obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d'accompagner celle-ci d'un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés. Il vise à inciter les personnes à se tourner vers des modes de transport actifs qui ont le double avantage d'être sans conséquence pour l'environnement et d'améliorer la santé en luttant contre la sédentarité, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, les jeunes Français sont trop sédentaires, avec un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans et les deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans qui passent plus de trois heures par jour devant un écran. S'agissant des adultes, 80 % sont également trop sédentaires. Cette proposition rejoint celle de Santé publique France, qui prévoit en 2019 de véhiculer un message simple incitant à « pratiquer des activités physiques dynamiques pendant au moins 30 minutes par jour

Il s'agit de créer une obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d'accompagner celle-ci d'un message en faveur des mobilités moins polluantes comme les mobilités actives, les transports en commun ou les mobilités partagées.

de loi qui nous semblait excellente : rendre obligatoire la promotion des mobilités actives dans chaque publicité pour la mobilité routière, à l'instar de la législation en vigueur relative à la publicité en faveur de produits alimentaires trop gras ou trop sucrés. En termes de santé publique, une telle démarche nous semble pertinente à double titre. D'une part, la mobilité routière est l'un des principaux facteurs de la pollution atmosphérique, qui tue chaque année 67 000 personnes, soit plus que le tabac, pour lequel, rappelons-le, la publicité est totalement interdite. D'autre part, selon certaines études, la sédentarité tue également plus que le tabac. Elle favorise le développement de facteurs de risques cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol trop élevé, l'obésité et tous les troubles musculo-squelettiques. Pour toutes ces raisons, il nous paraît cohérent d'obliger les publicités pour les voitures à faire figurer un message de prévention de santé publique enjoignant nos concitoyens à marcher ou à faire au moins trente minutes de vélo par jour. C'est aussi important que la consommation de cinq fruits et légumes par jour.

Cet amendement est construit sur le modèle des prescriptions déjà prévues par la loi à l'égard des publicités des industries de l'agroalimentaire et des spiritueux, qui doivent notamment communiquer sur la nécessité d'une alimentation saine ou sur les dangers de la consommation excessive d'alcool. De la même manière, nous proposons que les publicitaires de l'industrie automobile intègrent dans leurs annonces des messages en faveur des mobilités actives ou des alternatives à la voiture, comme l'usage des transports publics. Il s'agit non pas d'opposer frontalement mobilité active et mobilité automobile, mais au contraire d'insister sur leur caractère complémentaire, en sachant que l'essentiel des déplacements annuels des Français s'effectue dans un rayon strictement local.

voire d'une véritable incohérence : on prend ainsi prétexte de la sédentarité des jeunes enfants ou des heures passées par les adolescents devant des écrans pour justifier un message apposé sur des publicités pour la mobilité routière, qui s'adressent en principe à des personnes en âge d'acheter une voiture et de la conduire Pour lutter plus directement contre les écrans, peut-être vaudrait-il mieux cibler la publicité pour ces écrans eux-mêmes. J'ajoute que les messages sanitaires figurant sur les produits alimentaires recommandent déjà de pratiquer une activité physique régulière. Je suis par ailleurs très réservé à l'idée, au fond assez infantilisante, que les Français auraient besoin qu'on leur rappelle qu'il vaut mieux privilégier les transports en commun ou les mobilités propres ou partagées à l'usage de la voiture thermique. Ce serait du reste assez stigmatisant pour tous nos concitoyens, et ils sont nombreux, qui n'ont aujourd'hui pas d'autre solution pour se déplacer, sans parler du paradoxe qu'il y aurait pour des industriels à promouvoir leur produit tout en préconisant de ne pas l'utiliser ... Sur la forme, les insuffisances et les limites du dispositif proposé sont très nombreuses. On vise la mobilité routière, ce qui inclurait tous les véhicules circulant sur la voirie routière, qu'ils soient équipés ou non d'un moteur émettant ou non des gaz à effet de serre ou des polluants atmosphériques, ou encore qu'ils soient individuels ou collectifs., il conviendrait de viser la mobilité thermique individuelle- mais cela inclurait encore l'autopartage, qui doit au contraire être promu. Tous les messages publicitaires seraient concernés, et non uniquement ceux qui sont émis depuis et à destination du territoire national, dispositif que l'on serait bien en peine de mettre en oeuvre, notamment sur internet. Le champ des mobilités promues serait lui-même très difficile à établir inclurait-on, par exemple, dans les mobilités actives, l'usage des vélos à assistance électrique, qui consomment de l'énergie dont on pourrait se passer pour se déplacer à vélo- la meilleure énergie reste toujours celle que l'on ne consomme pas ? Dans les transports en commun, faudrait-il exclure les bus thermiques, ceux qui fonctionnent au GNV ou les hybrides ?

d'autant que le ministère de l'économie et des finances travaille plutôt dans le sens d'une réduction du nombre de mentions obligatoires dans les publicités. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Pascale Bories, pour explication de vote.

sociale. Je demande au Premier ministre, et non pas au rapporteur, d'en faire une cause nationale et de développer une campagne de communication nationale, non pas sur les véhicules,

mais je trouve que les supports de communication proposés ne sont pas assez ambitieux, donc je suivrai le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure. Le constat de la baisse de fréquentation des centres-villes est unanime. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déployé le plan « Action coeur de ville

La plupart des accidents en milieu urbain sont liés à la proximité des passages pour piétons, et ont pour cause une mauvaise visibilité à la fois pour les piétons, notamment les personnes âgées ou les enfants, et pour les conducteurs, qui sont gênés

L'augmentation de la mortalité des piétons impose des mesures fortes pour la sécurité des personnes vulnérables sur la chaussée. La visibilité des piétons est notamment susceptible d'être compromise lorsque des véhicules stationnent en amont des passages piétons. C'est ce qui avait conduit à retenir la mesure introduite par votre commission, mesdames, messieurs les sénateurs, lors du comité interministériel de la sécurité routière pour des aménagements neufs ou des réaménagements importants. Je suis défavorable à la suppression de cette disposition.

introduit en commission par le rapporteur, prévoit que seuls les vélos, vélos à assistance électrique et engins de déplacement personnel peuvent stationner sur les cinq mètres de chaussée précédant un passage pour piétons. Nous proposons d'étendre cette possibilité aux deux-roues à motorisation électrique, car ces véhicules offrent les mêmes garanties en matière de visibilité pour la traversée des piétons. La présence d'espaces de stationnement supplémentaires pour les deux-roues électriques permettra, en outre, d'encourager la transition vers des deux-roues à motorisation zéro émission et zéro bruit en ville. La parole

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous saluons la volonté des auteurs de ce texte de donner pour la première fois une définition juridique aux mobilités actives, mais nous souhaitons la compléter. Si leur caractère écologiquement vertueux a été mis en avant, il faut cependant souligner que ces mobilités favorisent aussi la santé publique. En effet, ces modes de déplacement quotidien, en

? Nous sommes tous d'accord pour dire que les mobilités actives, comme la marche ou le vélo, sont bénéfiques en termes de santé publique. C'est une évidence. Toutefois, l'ajout proposé par le biais de cet amendement n'est pas très précis, mes chers collègues, que les mobilités actives contribuent aux objectifs définis par le Haut Conseil de la santé publique, sans mentionner lesdits objectifs. Or certains de ces objectifs, qui touchent par exemple à l'organisation du système de santé, n'ont aucun lien avec les effets bénéfiques des mobilités actives. L'avis de la commission est défavorable.

monsieur Gontard. En l'état actuel du projet de loi, la section 1 ne comporte qu'une définition. Nous proposons d'y adjoindre un objectif de déploiement des mobilités actives par les autorités chargées de la politique des transports, dont la responsabilité est ainsi précisée. Cette disposition nous semble indispensable pour traduire dans les faits les objectifs de ce projet de loi et s'assurer qu'ils ne demeurent pas au stade de l'intention. En effet, si nous n'allons pas jusqu'à un droit à la mobilité active, il est néanmoins essentiel que son développement soit confié aux autorités organisatrices de transport. Malgré des politiques ambitieuses de construction d'infrastructures de transports en commun, la fracture territoriale ne s'est pas résorbée, à tel point qu'en 2018 plus de sept millions de personnes en âge de travailler, soit 20 % de la population active, rencontrent des difficultés pour se déplacer. Ces difficultés n'ont pas été résolues par les politiques menées jusqu'à ce jour, alors même que 85 % des Français résident à moins de cinq kilomètres d'un service public ou d'un mode de transport. La mobilité active, envisagée dans une perspective intermodale, est donc une réponse très concrète au besoin de mobilité de nos concitoyens.

Le développement des mobilités actives passe par des politiques concrètes, en matière notamment de développement des infrastructures cyclables et de lutte contre le vol des vélos. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La formule proposée par les auteurs de cet amendement est très générale. Elle n'a donc pas beaucoup de portée en tant que telle,

l'avis du Gouvernement ? Je partage bien sûr votre objectif, monsieur Gontard. C'est d'ailleurs pourquoi l'article 22 prévoit de créer dans le code des transports un titre spécifique dédié aux mobilités actives et à l'intermodalité. Il s'agit également de donner une définition des mobilités actives. Par ailleurs, le plan Vélo et mobilités actives, qui a été présenté par le Premier ministre en septembre dernier, intègre de nombreuses mesures sur l'éducation, les aménagements des infrastructures, la sécurité, la lutte contre le vol. vol. L'ajout que vous proposez ne me paraît pas nécessaire en droit. Toutefois, comme il confirme l'importance des mobilités actives, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

qui, pour certains, ont leur propre canal de distribution, sont pleinement engagés dans la réflexion sur un dispositif de marquage à la source internalisé, il est important de prévoir une date d'entrée en vigueur qui soit en phase avec les processus de fabrication déjà engagés. Nous proposons donc de reporter l'entrée en vigueur

en facilitant le démantèlement des réseaux de recel et de permettre la restitution des vélos. La plupart des acteurs ont d'ores et déjà commencé à s'adapter. Les travaux techniques s'inscrivent donc dans ce temps et permettent la mise en oeuvre de la mesure au 1 juillet 2020.

Il doit être économiquement et socialement efficient. Or le marquage représenterait une augmentation du prix sur les vélos enfants disproportionnée par rapport au prix de vente.

article prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine notamment les obligations faites aux vendeurs de vélos. La lutte contre le vol de vélos doit être une priorité, tant celui-ci représente un frein psychologique et économique au changement de mode de mobilité pour de nombreuses personnes. Cet amendement tend donc à préciser les contours du décret qui devra être pris. L'ensemble de la chaîne devant être mobilisé pour lutter efficacement, efficacement, il paraît nécessaire de préciser les différents acteurs chargés de la conception, de la gestion et de la maintenance du fichier national unique, ainsi que les modalités de financement.

l'amendement n° 987 rectifié. Le présent amendement vise à mieux encadrer le fichier national d'identification des cycles créé par l'article 22. En effet, la création d'un traitement automatisé à l'échelle nationale est toujours sensible en matière de libertés individuelles en plus, la gestion du futur fichier par des opérateurs ayant obtenu l'agrément de l'État est également susceptible de soulever des questions. Même si on ne peut que partager l'objectif de lutte contre le recel et le vol des cycles, il ne me semble pas raisonnable de renvoyer de manière aussi vague le règlement de la question et les conditions précises d'élaboration et d'administration du fichier. raison pour laquelle cet amendement a pour objet d'énumérer de façon plus claire les éléments qui devront être détaillés par décret.

de créer une procédure sécurisée pour l'identification des vélos, à l'image de ce qui existe déjà pour le marquage des mini-motos. En effet, l'identification de ces fait l'objet d'une procédure sécurisée grâce à un fichier géré par le ministère de l'intérieur. Ce fichier dispose d'un site internet dédié et opérationnel, qui délivre un numéro unique d'identification pour ce type de véhicules. Ainsi,

de préciser le contenu du décret d'application relatif à la mise en oeuvre du fichier des vélos identifiés, donnent à ce dernier une fonction supplémentaire, celle de recenser les lieux de survenance des vols de vélos.

Être l'objet d'un vol est très dissuasif puisqu'un quart des victimes ne rachètent pas de vélo. Afin de limiter le risque de vol et d'encourager les usagers à l'achat et à l'usage du vélo pour leurs déplacements quotidiens, notamment lorsqu'il s'agit de déplacements multimodaux combinant l'usage du vélo et celui des transports en commun, les gares et les pôles d'échanges multimodaux doivent comporter des emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos, et ce en nombre suffisant.

Ils doivent, de plus, être prévus en nombre suffisant, ce qui est rarement le cas à l'heure actuelle. La date du 1 janvier 2024 correspond à l'échéance fixée par le Gouvernement pour le plan Vélo, ainsi qu'à l'année où la France recevra les jeux Olympiques.

les vélos en fonction de la taille des gares et de la fréquentation. Il s'agit d'éviter de créer des obligations d'équipement dans des gares où les besoins ne sont pas forcément importants et de prévoir de tels équipements là où ils sont nécessaires. Nous avons laissé de la souplesse pour permettre une

l'amendement n° 863 rectifié. Cet amendement vise à équiper les stationnements sécurisés prévus par le présent projet de loi de prises de courant pour la recharge des batteries des cycles à pédalage assisté. L'autonomie de ces batteries varie en fonction de la capacité de ces dernières, du poids de l'usager, mais également de la durée d'emploi de l'assistance électrique. Après avoir parcouru un long trajet depuis chez soi, devoir recharger sa batterie sur son lieu de travail d'une autonomie suffisante pour le retour est un élément dissuasif de la pratique. Selon le lieu de travail, selon l'organisation de la journée ou des déplacements prévus, la charge de la batterie peut même être impossible. Cet aménagement contribuerait à une meilleure organisation pour les usagers. Équiper les parcs de prises de courant est un premier pas vers le changement de mobilité et inciterait nos concitoyens à se déplacer autrement. Je veux rappeler des chiffres cités précédemment : 35 % des déplacements en voiture

en fonction de la part modale du vélo sans pour autant pouvoir être inférieur à 1 % du trafic quotidien dans ladite gare. Les auteurs de l'amendement estiment que c'est à cette échelle, plus proche des réalités et avec une analyse plus fine du territoire, qu'il est pertinent d'agir, là où les caractéristiques des parkings peuvent être définies à l'échelon national. Il est proposé de fixer un nombre minimal

à M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions adoptées en commission relatives au stationnement des vélos dans les gares, enjeu clé de l'intermodalité. Le rapporteur avait alors refusé l'amendement que nous avions déposé, considérant qu'un taux de 2 % du trafic journalier pouvait représenter un nombre inconsidéré de stationnements dédiés aux vélos dans certaines gares très fréquentées. Il avait opportunément pris comme exemple le cas de la gare du Nord, la plus fréquentée du continent, pour nous opposer le chiffre de 14 500 places de stationnement consacrées au vélo, chiffre jugé parfaitement farfelu. En premier lieu, nous tenons à préciser que ce chiffre est en fait loin d'être déraisonnable pour un pays qui a pour ambition de développer le vélo. Ainsi, la gare d'Utrecht, aux Pays-Bas, vient d'achever un parking pour les vélos de 12 500 places. Ce parking étant largement insuffisant selon les usagers, la municipalité déploie un nouveau projet pour porter à 33 000 le nombre de places de stationnement sécurisées

Néanmoins, nous comprenons l'émoi de la RATP, la gare du Nord ne comptant quasiment pas une seule place de stationnement consacrée au vélo sécurisée. Elle part donc de très loin. Raison de plus pour inscrire dans la loi un objectif digne de ce nom

Cet amendement vise à assurer un seuil de places suffisant pour le stationnement sécurisé de vélos, qui serait indexé sur la fréquentation des usagers dans les gares et les pôles d'échanges multimodaux.

de contractualisation avec le gestionnaire des gares. Si ce dernier s'opposait au nombre retenu par l'AOM, de quel recours disposerait-elle pour le contraindre à s'exécuter ? Il convient donc d'en rester à la rédaction de l'article, qui prévoit une obligation d'équipement des gares de niveau législatif,

l'autorité organisatrice ne pourra pas forcément imposer des obligations différentes à un gestionnaire de pôle d'échanges ou de gare. On fragiliserait le dispositif en ne s'appuyant pas sur un décret, comme cela est proposé actuellement.

pour trouver des emplacements de substitution pour les vélos lorsque leurs emprises ne suffisent pas. Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 inclut les abords des gares dans les zones concernées. Or ni la SNCF ni la RATP ne sont gestionnaires ou propriétaires de voiries aux abords de leurs infrastructures. Aménager des emplacements pour les vélos aux abords des gares n'est donc pas une question qui les

de l'obligation en tenant compte des besoins constatés selon notamment qu'il s'agit d'un déplacement de proximité ou de longue distance, ainsi que des caractéristiques des matériels concernés.

envisagée de la façon la plus large possible. Les cyclistes ont une forte préférence pour le train quand ils rejoignent un itinéraire ou en repartent. Une intermodalité embarquée est donc capitale pour proposer une alternative de mobilité crédible. Les trois amendements

Cependant, l'absence de stationnements sécurisés hors agglomération et la nécessité de disposer d'un vélo au départ et à l'arrivée d'un trajet intermodal sont des freins à son développement. Aussi proposons-nous de généraliser une pratique déjà courante dans plusieurs départements et régions de France, et dans la plupart de nos pays voisins les cars neufs sur les lignes régulières ou saisonnières, hors services urbains bien sûr, sont équipés d'un système homologué de chargement de cinq vélos non démontés, afin de faciliter les intermodalités. Quel

je veux souligner qu'il n'existe pas aujourd'hui, en dehors du transport en soute, de dispositif homologué pour transporter des vélos par autocar. L'emport des vélos à bord de ces véhicules est soumis à des contraintes fortes, relevant à la fois de la sécurité routière- les systèmes de transport de vélos doivent être montés à l'arrière, sous peine de contrevenir à l'article R. 312-22 du code de la route, et cela sans bloquer la fenêtre arrière qui, selon les véhicules, peut constituer une issue de secours de secours -et de difficultés techniques, puisque la longueur des véhicules est normée par des réglementations internationales- c'est pourquoi l'ajout de dispositifs permettant l'emport extérieur de vélos n'est pas possible

92 % des cyclistes confient craindre pour la sécurité de leur monture. Les gares et les pôles d'échanges multimodaux ne peuvent être les seuls emplacements ciblés par le dispositif de sécurisation des stationnements pour les vélos en ville. en ville. Cet amendement vise donc à accélérer la création de places de stationnement sécurisées pour les vélos dans les parcs de stationnement existants lors de la réalisation de travaux dans des bâtiments à usage industriel ou tertiaire ou accueillant un service public ou commercial. ces mesures sont inscrites au point 15 du plan Vélo annoncé par le Premier ministre. Quel

l'échelon réglementaire, préciser les dispositions qui devront être prises, avec à la fois des installations très sécurisées pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, des locaux clos et couverts dotés de systèmes de fermeture sécurisée, et, sans doute, des mesures moins contraignantes pour les parcs annexes aux bâtiments de service public et pour les ensembles commerciaux, dans lesquels pourraient être prévus des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher des vélos.

à M. Laurent Lafon. On sait que le stationnement des vélos en ville pose des problèmes de sécurité pour les propriétaires de vélos ; il pose aussi des problèmes de gestion de l'espace public pour les responsables des communes.

lorsqu'un PLU prévoit, pour les immeubles d'habitation et de bureaux, des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, les obligations relatives au stationnement des vélos soient renforcées. Sensibles à l'argument avancé par M. le rapporteur, en commission, concernant notre première proposition d'amendement-

fréquemment, les PLU définissent les obligations en matière de places de stationnement pour les véhicules par nombre d'emplacements à réaliser. Or une place de stationnement pour les véhicules motorisés peut accueillir au moins cinq places de stationnement pour les vélos. En imposant une équivalence, le nombre de places dédiées aux vélos serait dans certains cas divisé par cinq.

n° 43 rectifié . Dans le droit fil du bouleversement majeur que nous attendons tous concernant les petits et les micro-déplacements, cet amendement vise à développer le réflexe vélo chez les plus jeunes, afin d'inscrire durablement le vélo dans les habitudes, comme un mode de déplacement régulier, conformément, d'ailleurs, à la mesure n° 10 du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018. L'objectif de cette mesure est d'accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Cela signifie, pour les enfants, généraliser le « savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies, et qui viendrait s'ajouter aux autres savoirs essentiels que les élèves doivent maîtriser à leur entrée en sixième, le « savoir nager » par exemple, et ce afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie à vélo en vue de l'entrée au collège. Les établissements d'enseignement du premier degré devront apprendre aux élèves à se déplacer à vélo de manière autonome et sécurisée dans des conditions de circulation réelles. Ainsi, dès leur entrée dans le secondaire, l'ensemble des élèves pourront-ils utiliser le vélo pour tout ou partie de leurs trajets quotidiens vers le collège, selon l'éloignement de celui-ci. Cette mesure aura également des effets positifs en matière de santé publique, puisque les jeunes auront ainsi une occasion supplémentaire de pratiquer une activité physique, ce qui, comme chacun sait, est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour lutter contre la sédentarité et contre l'obésité.

Nous pensons, pour notre part, que l'école doit accompagner les familles pour favoriser cet apprentissage par tous les élèves. Trop de nos concitoyens, aujourd'hui, n'utilisent pas le vélo ; en effet, son usage et son apprentissage ne sont pas répandus dans tous les milieux sociaux, soit pour des raisons financières, soit parce que certains parents ne maîtrisent pas eux-mêmes la technique du vélo. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'envisager seulement l'apprentissage du vélo dans un jardin ou un chemin : il s'agit bien d'un apprentissage de la route, et donc, notamment, de notions du code de la route, afin de former de futurs cyclistes responsables et prudents. C'est justement le rôle de l'école d'apporter une base commune de savoir à tous nos futurs citoyens, et le « savoir rouler doit en faire partie, car nous savons que, en tant que moyen de transport décarboné, le vélo occupera une place toujours plus importante dans la mobilité de demain. Nous souhaitons donc que, au même titre que le « savoir nager », l'école délivre l'attestation d'un « savoir rouler ».

à se plaindre de l'état de santé de notre jeunesse, constater qu'aujourd'hui les jeunes passent plus de temps assis devant un écran qu'à faire une activité physique,

dans des conditions optimales de sécurité. C'est bien dans ce sens qu'a été élaboré un programme d'apprentissage du « savoir rouler à vélo » à destination des enfants de six à onze ans. Cet engagement du Gouvernement est à la confluence de différentes politiques, de sécurité routière, de santé, de mobilité et de sport. Sous l'impulsion du ministère des sports, en liaison avec les ministères des transports, de l'intérieur et de l'éducation nationale et de la jeunesse, tous les acteurs

de pratiquer quotidiennement une activité physique bonne pour la santé ; il doit permettre également de promouvoir des déplacements à moindre empreinte carbone. Le lancement de ce programme est prévu en avril, il sera déployé sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. L'objectif est bien de généraliser l'apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l'ensemble des enfants avant l'entrée au collège,

ou encore la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes, non seulement les ministères que j'ai mentionnés, mais aussi tout l'écosystème du vélo, le monde associatif, éducatif et sportif.

j'ai construit un équipement sportif intégré, un bassin d'initiation à la natation, une salle de sport et j'ai mis en place un parcours de santé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand j'entends qu'on pourrait substituer au sport à l'école

se mêle. Un plan pour mettre en oeuvre ce « savoir rouler » et veiller à ce que l'ensemble des jeunes entrant en sixième à partir de 2022

dans le cadre des horaires des établissements. Or le plan qui est élaboré depuis plusieurs mois avec tous les partenaires, notamment les fédérations sportives et les associations de sécurité routière, prévoit que l'enseignement peut aussi s'effectuer sur les temps périscolaire ou extrascolaire.

Cette mobilité est d'autant plus attractive que, selon France Stratégie, les prix des voyages en autocar sont dans la plupart des cas inférieurs à ceux des covoiturages et toujours inférieurs à ceux du train. Toutefois, les capacités d'accueil des agglomérations restent insuffisantes, et l'accès des cars est difficile dans certaines villes. Il est donc nécessaire que des gares routières soient aménagées ou rénovées et qu'elles s'intègrent- c'est le sens de cet amendement -dans une réflexion multimodale plus large. Car les pôles d'échanges multimodaux constituent un maillon essentiel de l'attractivité des réseaux de transport. Ils doivent être développés, afin d'assurer un maillage territorial cohérent, au service des besoins de mobilité de nos concitoyens. La création d'un nombre suffisant de places de stationnement d'autocars, que j'appelle de mes voeux, pourrait ainsi se faire en fonction du flux de passagers, afin d'offrir à ces derniers des conditions de confort et de sécurité supérieures et de leur garantir l'ensemble des services de transport dont ils ont besoin. La parole

pour lesquels il constitue parfois l'unique moyen de transport public. Toutefois, de nombreux accidents surviennent lors de la montée et de la descente des véhicules. Afin d'éviter cela, je propose de pré-signaler les arrêts hors agglomération dédiés au transport scolaire.

Une telle préoccupation est légitime, mais le moyen choisi est peut-être disproportionné. En effet, dans les territoires ruraux en particulier, les arrêts sont amenés à changer régulièrement au gré

de ces amendements identiques souhaitent que les arrêts hors agglomération dédiés au transport scolaire soient pré-signalés. Je suis évidemment particulièrement attentive à la sécurité des enfants et du transport scolaire. Aujourd'hui, la réglementation prévoit que la signalisation et la pré-signalisation sont facultatives. Il est proposé de systématiser cette pré-signalisation. Je suis tout à fait favorable à ce que nous examinions cette disposition, en liaison avec les gestionnaires routiers.

jouent un rôle fondamental dans le développement de la marche et du vélo. Le code de la route a déjà évolué, et il évoluera à la suite des décisions prises dans le cadre du plan Vélo et mobilités actives, avec l'introduction du principe de prudence à l'égard de l'usager vulnérable, la redéfinition de certaines zones de circulation apaisée, la généralisation des doubles sens cyclables dans les zones 30 et les zones de rencontre, le renforcement de la priorité du piéton lors d'une traversée de chaussée, la création du panneau cédez-le-passage cycliste au feu rouge, la création du stationnement très gênant, la sécurisation juridique de la généralisation du 30 kilomètres par heure en ville, la modification du code de la route pour permettre aux automobilistes de chevaucher la ligne blanche lorsqu'ils dépassent un cycliste, la généralisation des sas vélos et l'encadrement des nouveaux modes de déplacement, notamment des engins de déplacement personnel.

pas toujours le code de la route. Nous invitons par conséquent le Gouvernement, très attaché à la sécurité routière, à réfléchir à la mise en oeuvre d'un dispositif peu onéreux, mais qui sauverait de nombreuses vies. Quel

C'est pourquoi nous avons décidé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité de ces usagers dans le cadre du plan Vélo et mobilités actives. Je veux notamment évoquer la généralisation, dont nous venons de débattre,

en particulier dans les zones urbaines : de 300 000 à 500 000 vélos sont volés chaque année. L'objectif du Gouvernement de porter à 9 % d'ici à 2024 la part des déplacements faits en vélo pour dépasser la moyenne européenne de 7 % ne pourra pas être atteint sans la mise en place d'une politique forte de lutte contre le vol et contre les détériorations. Les gares et les pôles d'échanges multimodaux ne peuvent pas être les seuls emplacements ciblés par le dispositif de sécurisation des stationnements pour les vélos en ville si l'on veut que les usagers prennent leur vélo dans des conditions sécurisées depuis leur domicile jusqu'à leur lieu de travail. Cet amendement vise donc à accélérer la sécurisation des stationnements pour vélos, qui sont déjà obligatoires lors de la construction de bâtiments accueillant un service public ou de bâtiments commerciaux ou accueillant un établissement cinématographique. Une telle mesure s'inscrit en parfaite cohérence avec l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit l'aménagement de stationnements sécurisés lors de la construction de bâtiments d'habitation ou de bâtiments à usage industriel ou tertiaire. La parole

Quel est l'avis de la commission ? accueillant un service public ou constituant un ensemble commercial doivent être sécurisés, comme c'est le cas actuellement s'agissant des bâtiments d'habitation ou à usage industriel ou tertiaire. La rédaction proposée par le sous-amendement du Gouvernement, qui vise à compléter ces amendements, afin que la sécurisation des places dédiées aux vélos soit proportionnée au risque, est pertinente. C'est pourquoi la commission est favorable

Cet amendement n'ajoute pas de contrainte pour les collectivités. Il vise à simplifier la vie dans les copropriétés : lorsqu'un copropriétaire s'oppose

l'amendement n° 362. Cet amendement s'explique de lui-même : il s'agit d'étendre les dispositifs de l'article 24 du présent projet de loi, relatif aux bornes de recharge des véhicules électriques, aux stationnements sécurisés pour les vélos. En effet, l'article 24 prévoit, quand les conditions le permettent, qu'un propriétaire ou une copropriété ne peut pas s'opposer à l'installation à ses frais par un copropriétaire ou un locataire d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Nous proposons d'élargir cette mesure de bon sens aux stationnements pour vélos sécurisés, qui sont des investissements beaucoup moins lourds et onéreux. Nous y adjoignons également une clause de retrait.

dite loi ÉLAN, a permis de travailler sur les questions relatives aux copropriétés. L'usage des parties communes d'une copropriété est normalement soumis à un accord en assemblée générale. Permettre à un copropriétaire ou à un locataire d'installer dans ces parties communes des équipements pour vélos sans l'accord des autres copropriétaires pourrait être de nature à multiplier les conflits au sein des

ne sont pas de même nature que ceux qui sont dits d'« amélioration », tels que l'aménagement d'emplacements de stationnement déjà existants dans un parking.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de la politique d'identification, une évaluation de l'efficacité de cette politique, en lien avec le nombre d'infractions recensées et les améliorations éventuelles à y apporter. Je partage souvent la réticence du Sénat à l'égard de nouveaux rapports.

Même avis. Une convention triennale de partenariat a été conclue entre la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, et les services de police et de gendarmerie sur le sujet très important de la prévention

de renforcer la lutte contre le vol de vélos et le recel grâce au développement de garages sécurisés et à la mise en place d'un marquage pour la mise en vente.

vise à rendre obligatoire pour les régions la mise en place d'un schéma régional des véloroutes avant le 31 décembre 2025. L'enjeu économique de ces schémas est très important puisqu'en 2014 le tourisme à vélo représentait 9,2 millions de séjours, en comptant les 25 % de touristes étrangers qui choisissent ce mode de déplacement. C'est un chiffre d'affaires global estimé à 2 milliards d'euros, et l'une des filières les plus dynamiques du marché touristique français. De plus, les grands itinéraires cyclables ont un rôle structurant pour les territoires et sont majoritairement empruntés par les usagers quotidiens pour leurs déplacements utilitaires. L'amendement tend en outre à donner une définition légale contraignante des véloroutes, qui, contrairement aux voies vertes, ne font pas l'objet d'une telle définition aujourd'hui. Par ailleurs, il a pour objet de supprimer le décret d'application prévu pour le schéma national des véloroutes et voies vertes puisque les dispositions législatives du nouvel article L. 1212-3-4 du code des transports sont suffisamment précises.

les documents de planification de niveau infrarégional pour tout ce qui concerne la mobilité. Le schéma national et les schémas régionaux des véloroutes constituant l'armature principale du réseau cyclable français, il semble donc opportun d'introduire ces schémas régionaux dans les Sraddet. Quel

Il peut s'agir d'itinéraires empruntant des voiries nationales, départementales, communales, des chemins ruraux ou forestiers, des chemins de halage, ou encore des voies vertes, et le statut de ces différentes voies varie beaucoup. Compte tenu de cette hétérogénéité, il ne paraît pas opportun de figer dans la loi une définition des véloroutes, au risque de ne pas être suffisamment exhaustif.

L'enjeu économique de ces schémas est très important puisqu'en 2014 le tourisme à vélo représentait 9,2 millions de séjours, en comptant les 25 % de touristes étrangers qui choisissent ce mode de déplacement. C'est un chiffre d'affaires global estimé à 2 milliards d'euros, et l'une des filières les plus dynamiques du marché touristique français. En outre, les grands itinéraires cyclables ont un rôle structurant pour les territoires et sont majoritairement empruntés par des usagers quotidiens pour leurs déplacements réguliers. Enfin, cet amendement tend à donner une définition légale contraignante des véloroutes, qui, contrairement aux voies vertes, ne font pas l'objet d'une telle définition. Quel est l'avis de la commission ? Ma position Ma position sera de simplification. Ces amendements paraissent satisfaits par l'article 22 que nous avons introduit en commission, lequel prévoit que les Sraddet devront identifier les itinéraires

rectifié . L'existence de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, depuis 1996, a permis la création d'un grand nombre d'itinéraires cyclables. Néanmoins, la rédaction actuelle de cet article a donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de vingt ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d'améliorer le dispositif existant. Cet amendement vise tout d'abord à élargir aux voies interurbaines l'obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu'une portion de voirie routière est réalisée ou rénovée. en plus de cyclistes souhaitent se déplacer en vélo entre les agglomérations dans des conditions sécurisées. Or la voirie départementale entre les agglomérations est souvent trop dangereuse pour eux. Des itinéraires sécurisés sont donc souhaitables. également que les intérêts des cyclistes soient pris en compte lorsque la voirie urbaine et interurbaine fait l'objet d'une création ou d'une rénovation. Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d'itinéraires cyclables entre agglomérations. J'ajoute qu'il convient de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu'il soit bien clair, comme l'a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l'aménagement cyclable qui doit être mis en oeuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée. En outre, la possibilité actuelle de réaliser un simple marquage au sol a permis, dans certains cas, de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d'ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois très dangereuses. Il convient dès lors de corriger ce point en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l'option choisie, sécurisés. De même, une application parfois quelque peu négligente de l'article L. 228-2 du code de l'environnement a conduit à la création d'itinéraires cyclables en « patchwork », c'est-à-dire non continus ou interrompus, spécialement au niveau des carrefours, où le risque d'accident est justement le plus grand pour les cyclistes.

L'allure actuelle de patchwork, qui vient d'être rappelée, de notre réseau de pistes cyclables n'est pas à la hauteur des objectifs ambitieux du passage de 3 % à 9 % de la part modale du vélo qui ont été fixés par le plan Vélo. nous félicitons, en ce sens, de l'adoption en commission de l'amendement 45 rectifié, qui permet d'étendre les obligations de construction d'aménagements cyclables, prévues par la loi sur l'air Cependant, il nous paraît que l'article L. 228-2 du code de l'environnement mérite une nouvelle rédaction d'ensemble. En effet, son interprétation par les juridictions administratives déforme souvent l'esprit initial de la loi. La pondération en fonction des besoins et contraintes de la circulation doit s'appliquer au choix du type d'infrastructures cyclables adaptées, et non à la question de la pertinence ou pas d'installer une ou pas d'installer une infrastructure cyclable selon ces contraintes. Pour en finir avec cette erreur d'interprétation, nous proposons cette rédaction qui nous paraît plus limpide. Nous proposons également d'inscrire un critère de continuité et de sécurité des itinéraires cyclables, indispensable pour garantir une pratique confortable limiter les risques d'accident, notamment aux carrefours. Même si, en raison des contraintes de la circulation, l'infrastructure choisie est un marquage au sol, celui-ci doit être conçu avec l'objectif d'assurer la sécurité des cyclistes ; il faut ainsi qu'il soit d'une largeur suffisante, avec un revêtement de bonne qualité et des aménagements spécifiques aux intersections. Ces critères de continuité et de sécurité sont essentiels à l'adoption d'une pratique quotidienne du vélo. Enfin, nous proposons de supprimer de l'article la mention des PDU, qui n'apporte rien d'autre que de la confusion. La

Or l'aménagement des pistes cyclables doit répondre à des principes rigoureux de conception et être très adapté au contexte local,

entre le gestionnaire de la voirie et la ou les autorités organisatrices de la mobilité, afin d'analyser la sécurité du projet, sa pertinence par rapport aux objectifs d'aménagement, son coût et le respect des schémas déjà arrêtés.

Par conséquent, il convient plutôt de retenir la solution proposée au travers de l'amendement n° 296 rectifié de M. Fouché, lequel prévoit que les gestionnaires de voirie soient tenus, lors de la réalisation de l'aménagement de voies interurbaines, d'évaluer le besoin de réaliser des itinéraires cyclables,